À seize heures trente, le soir et la nuit : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

peut être bénéficiaire net des écocontributions aux éco-organismes lorsqu'il s'inscrit dans des pratiques particulièrement vertueuses. L'écocontribution est la contrepartie financière annuelle versée par une entreprise à un éco-organisme agréé pour la prise en charge de l'élimination des déchets produits par ses activités, en vertu d'une filière REP. La filière emballages est particulièrement concernée par cet article. Actuellement, la très grande majorité des producteurs contribuent à l'un des trois éco-organismes agréés. Ces derniers reversent reversent les contributions perçues sous forme de soutien aux collectivités pour le financement du dispositif de collecte séparée, du tri et du recyclage des déchets d'emballages ménagers. Le tri à la source des déchets d'emballages ménagers est pratiqué par une très grande majorité de Français. Cependant, un effort reste à faire sur la qualité du geste de tri pour maîtriser les coûts de la filière et faciliter le recyclage. Quel est l'avis de la commission ? Favorable.

en compagnie du maire et des élus, que j'ai constaté que nos entreprises avaient de la ressource : nous sommes en train de constituer un écosystème industriel pertinent à l'échelle du département, allant de la production au recyclage, en passant par l'utilisation. Au-delà de la question du PS et du PSE, c'est toute la filière agroalimentaire qui s'interroge. Les emballages à base de polymère de polymère styrénique sont indispensables pour la conservation et la production de nombreux produits, notamment des produits d'origine animale tels que le poisson ou la viande. La filière du transport de marchandises, lequel a explosé lors du confinement, est tributaire des emballages de protection. Nos collègues de la commission ont modifié le texte initial afin d'exclure de l'interdiction les polymères recyclables.

Cette interdiction introduite dans le projet de loi, sans étude d'impact, mettrait un coup d'arrêt à l'ensemble des initiatives et enverrait un signal particulièrement négatif à nos industriels.

Il ne nous paraît pas opportun, comme le propose la commission, de créer une exception à l'interdiction des polymères ou des copolymères styréniques, plus connus sous leur nom d'usage de polystyrènes.

Dans la logique de cet objectif, l'Assemblée nationale propose d'interdire les emballages en polystyrène en 2025. En effet, le styrène, qui est utilisé dans la fabrication des polystyrènes, est hautement toxique

ce stade. Les plastiques styréniques nuisent au recyclage et représentent 42 % des plastiques incinérés. Ce n'est pas rendre service aux industriels que de créer cette exception pour des polystyrènes potentiellement

la commission ? La suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale concernant les emballages en polystyrène n'est pas opportune. Il nous a semblé plus sécurisant de trouver une solution équilibrée. est le sens de l'amendement que nous avons adopté en commission, visant à restreindre l'interdiction aux seuls emballages en polystyrène non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage à compter du 1 janvier 2025.

les objectifs européens de recyclage et grèvent notre bilan carbone. À l'heure où nous avons voté la sortie du plastique à usage unique dans la loi anti-gaspillage d'ici à 2040 et où nous avons fixé l'objectif de tendre vers 100 % de plastique recyclé d'ici au 1 janvier 2025, il est indispensable que les résines employées soient recyclables et disposent d'une filière de recyclage opérationnelle. Dans le cadre du pacte national sur les emballages plastiques, qui réunit des producteurs, des distributeurs, des et le ministère de la transition écologique autour d'engagements volontaires, certaines marques et des distributeurs de produits frais se sont saisis de ce sujet et ont appelé à une décision rapide des signataires concernés pour mettre fin à l'utilisation du polystyrène dans les emballages. L'Assemblée nationale s'est, elle aussi, saisie de cette question en votant-Mme la rapporteure l'a dit -l'interdiction des emballages en polystyrène en 2025. Le travail en commission, au Sénat, a cherché à rendre plus opérationnelle la mesure en la ciblant sur des emballages non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage. Dans ce contexte, les acteurs de la filière industrielle du polystyrène m'ont transmis, hier, une charte visant à réduire l'impact sur l'environnement des emballages qu'ils produisent, par laquelle ils s'engagent à développer une nouvelle filière de recyclage capable de produire une matière recyclée, avec retour au contact alimentaire : elle permettrait le recyclage effectif de 100 % des emballages en polystyrène collectés et triés en France en 2025. Le développement de cette filière s'appuiera sur des pilotes puis, dès 2023, sur des usines industrielles portées par Michelin, Ineos et Total.

La disposition votée en commission, au Sénat, me semble offrir un cadre approprié à l'engagement des acteurs de la filière du polystyrène. En complément, j'utiliserai le levier réglementaire relatif à la filière REP emballages, pour définir plus précisément la notion d'emballage recyclable et fixer des objectifs d'incorporation de matières recyclées. La filière REP emballages accompagnera aussi ces engagements grâce à un système de primes et de pénalités, renforcé dans le cadre de la loi de la loi anti-gaspillage. Cette dernière prévoit qu'un arrêté fixe, pour 2022, une pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage. Le polystyrène est par ailleurs, comme d'autres résines, concerné par le dispositif de bonus à l'incorporation de plastique recyclé dans des emballages, mis en place cette année. C'est pourquoi il ne me semble pertinent ni de revenir aux dispositions

issus de la vente à emporter et de la restauration livrée ; 85 % estimaient nécessaire de mieux lutter contre ces déchets. Le présent amendement vise à répondre à cette préoccupation en prévoyant que, à compter du 1 janvier 2025,

prévoit : « À compter du 1 janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter sont tenus de proposer au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. Même si une utilisation raisonnée des emballages en plastique à usage unique reste un objectif pour le respect de l'environnement, il est important de soutenir l'ensemble des solutions innovantes sur lesquelles les industriels de l'emballage travaillent déjà depuis quelques années. Cet amendement vise donc, aux côtés des solutions de réemploi ou d'utilisation d'emballages biosourcés, à inclure les emballages recyclables s'inscrivant dans des filières de recyclage opérationnelles, afin de poursuivre, dans la continuité

Si le papier et le carton qui composent les contenants alimentaires sont toujours recyclables et biosourcés, seuls certains plastiques utilisés pour les contenants alimentaires sont recyclables.

peuvent parfois être parfaitement recyclables, notamment en boucle fermée. À l'inverse, certaines matières biosourcées recyclables peuvent avoir un impact environnemental négatif, surtout lorsqu'elles perturbent le recyclage d'autres matériaux ou se retrouvent dans l'environnement. L'amendement

Notons qu'une telle pratique a déjà cours pour les bouteilles, mais reste limitée aux entreprises historiques faisant du réemploi. En Alsace, le format VK Alsace est déjà utilisé par deux marques : Meteor et Kronenbourg.

des consommateurs pour l'accès à des produits consignés réemployés, tout reste à faire. Les formats d'emballages réemployables n'existent pas encore. Inciter les producteurs à définir dès maintenant des gammes standardisées et limitées en nombre permettrait le développement rapide du réemploi et un gain environnemental maximal la massification des flux logistiques.

L'alinéa 3 de l'article 11 , qui a été introduit en commission, prévoit une expérimentation visant à faire obligation aux plateformes de vente en ligne de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné.

Mme la rapporteure, tend à décaler l'adoption du dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre après la publication de l'évaluation conduite par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation.

les enjeux de traçabilité ni la sécurité des consommateurs. Une consigne obligatoire va à l'encontre d'une filière solide, fleuron de nos exportations et de l'attractivité de nos territoires. Nous aurons l'occasion d'y revenir en présentant nos amendements, mais ne conviendrait-il pas de laisser les producteurs s'organiser et faire le choix de la consigne pour réemploi si elle est efficiente d'un point de vue économique et environnemental ? Madame la ministre, madame la rapporteure, essayez d'entendre les inquiétudes de la filière. Comment pouvons-nous imaginer consigner une nouvelle fois

Nous devons réduire nos déchets. Nous devons réutiliser tout ce qui peut l'être. Nous devons recycler autant que possible. Une bouteille en verre peut être réutilisée jusqu'à cinquante fois. Selon l'Ademe, la consigne permettrait d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie.

d'instituer un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Je m'interroge de manière générale sur le nombre d'observatoires, commissions et instances consultatives en France. Nous devenons les champions du monde en la matière. En 2020, on en comptait 387. Pour lutter contre le réchauffement climatique, on crée parfois paradoxalement des usines à gaz ! Un jour, on finira par créer un observatoire des observatoires

présidée par un Girondin -estimait qu'il était possible d'atteindre l'objectif de 90 % de collecte de bouteilles en verre en 2029 sans recourir à la consigne. Elle a pointé des pistes d'amélioration, comme le renforcement de la tarification incitative, la densification des points d'apport de proximité ou encore la mise en place d'un dispositif de contrôle du geste de tri. La solution repose sur la combinaison de ces différents leviers, auxquels peut s'ajouter un dispositif de consigne qui doit être volontaire. En effet, les bénéfices environnementaux d'une généralisation nationale d'un dispositif de consigne pour réemploi ne vont pas de soi.

encore en France -, le bilan environnemental est négatif. Or la France ne compte pas ou peu de bassins de consommation exclusivement régionaux. Les transports des bouteilles en verre vides à travers l'ensemble des territoires pourraient donc avoir un lourd impact environnemental. Des initiatives en matière de consigne naissent à l'échelon local sur la base du volontariat, y compris au sein de la filière viticole, très volontaire en la matière- je puis vous l'assurer -, lorsque le dispositif est adapté au regard de la demande et n'implique pas de transport de bouteilles vides sur des longues distances. Laissons aux producteurs la possibilité de s'adapter au contexte local sans leur imposer une obligation contre-productive du point de vue environnemental. Or la rédaction issue des travaux de la commission, qui prévoit qui prévoit la mise en place d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, rendrait le dispositif

! Cet amendement vise donc à revenir à l'équilibre trouvé par l'Assemblée nationale en supprimant cette trajectoire et en précisant le caractère volontaire du dispositif de consigne pour réemploi lorsque le bilan environnemental, économique et social global est positif, comme il l'est aujourd'hui. Très bien

alcooliques de la définition par décret d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Le réemploi du verre est principalement effectué les dispositifs de consigne et de vrac. Il est reconnu que, pour les bouteilles en verre destinées à contenir des boissons alcoolisées, soit près de 90 %, les possibilités de vente en vrac sont limitées et risquent de rendre le dispositif inopérant. La mise en place du dispositif de consigne pour réemploi doit être envisagée à l'aune de sa pertinence environnementale.

vise à supprimer la définition par décret d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire existe déjà dans les textes. En effet, l'article 67 de la loi

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a intégré, au sein de l'article 12, la définition par décret d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ce faisant, la généralisation de la consigne pour réemploi a désormais valeur contraignante. Comme je l'ai expliqué précédemment, la consigne pour réemploi est un dispositif inadapté aux besoins du secteur de la vigne et du vin. L'impact environnemental d'une telle mesure généralisée à l'échelle nationale est très incertain et potentiellement délétère. Il est indispensable de conserver le caractère volontaire du dispositif pour tenir compte des situations et des contextes au cas par cas et laisser les initiatives émerger.

ce qui me paraît préférable. Au demeurant, la pertinence environnementale et économique de la consigne pour réemploi des emballages en verre doit faire l'objet d'une évaluation avant le 1 janvier 2023- c'est demain. Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement. Cela ne signifie pas que la filière ne fait pas d'efforts.

Il nous paraît logique d'attendre les résultats de l'évaluation qui doit être menée d'ici au 1 janvier 2023 avant de statuer sur le réemploi des contenants en verre.

Comprenne qui pourra le raisonnement juridique subtil amenant à considérer l'absence de lien direct avec l'objet du projet de loi ... Pour tenir l'objectif de 2040, et l'objectif écologiste de 2030, il est indispensable de déployer la vente sans emballage et les emballages réemployables.

en 2030. Nous sommes lucides sur la hauteur des marches à gravir. Vous l'aurez noté, nous avons repoussé les échéances à un horizon ambitieux, donc atteignable. Ces objectifs s'inscrivent naturellement dans le mécanisme de la responsabilité élargie du producteur. Cela a également pour effet d'harmoniser les objectifs de réemploi pour l'ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers, qui souffrent aujourd'hui de nombreuses disparités. Ils ont également vocation à être retranscrits sous forme d'objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières REP des emballages ménagers et professionnels. L'amendement n° 300 rectifié,

et de 10 % en 2027. Le manque d'uniformité des objectifs, qui diffèrent en fonction des matériaux concernés, et l'absence de contraintes freinent les progrès en la matière. Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l'ensemble des matériaux de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et à les intégrer au sein des cahiers des charges des filières REP des emballages ménagers et professionnels, afin de les rendre plus contraignants, et donc d'assurer leur effectivité.

à mettre sur le marché devra être pris après la publication de l'évaluation du dispositif de consigne pour réemploi par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation. Celle-ci doit être effectuée avant le 1 janvier 2023.

Cet amendement de repli vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Le réemploi du verre est principalement effectué les dispositifs de consigne et de vrac. Il est reconnu que, pour les bouteilles en verre destinées à contenir des boissons alcoolisées, soit près de 90 %, les possibilités de vente en vrac sont limitées et risquent de rendre le dispositif inopérant.

Cela a été souligné, le réemploi du verre s'effectue principalement les dispositifs de consigne et de vrac. L'article 12 tel qu'issu des travaux de la commission dispose justement qu'une évaluation d'un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1 janvier 2023 par l'observatoire du réemploi de la réutilisation. Elle doit attester de sa pertinence environnementale et économique. Cela montre bien que l'intérêt du dispositif n'est pas encore assuré, d'autant que l'Ademe doit mener des travaux complémentaires. Plus encore, plus de 90 % des emballages en verre sont destinés à contenir des boissons alcoolisées, pour lesquelles le réemploi, déjà possible sous forme volontaire, n'offre que des avantages très limités compte tenu des enjeux de préservation de la qualité et de distance entre les lieux de production et les lieux de consommation.

Dès lors, et par cohérence, l'observatoire pourrait être chargé du suivi des informations et des études liées à la réparation, de l'impact du fonds de réparation sur le nombre de réparations effectivement réalisées,

plus de 90 % des 1 800 élus locaux qui ont répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi Climat et résilience estiment pertinent

verre soit réalisée avant 2023. En permettant d'identifier plus finement les secteurs et les emballages qui devront faire l'objet d'un dispositif de consigne, cette évaluation devrait permettre d'accompagner la montée en puissance du réemploi. L'amendement adopté en commission vise par ailleurs la définition par décret d'une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Il s'agit là de répondre à la demande forte de nos élus locaux en faveur du développement du réemploi du verre, tout en donnant de la visibilité aux metteurs sur le marché et en permettant un développement différencié selon les filières.

visant à préciser que le décret définissant la trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France ne pourra être pris qu'après l'évaluation environnementale et économique réalisée par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation.

Je suis également défavorable aux amendements 771 rectifié et 300 rectifié, qui visent à accroître les objectifs de mise sur le marché d'emballages réemployés. La loi AGEC prévoit déjà des objectifs de mise sur le marché d'emballages réemployés 5 % en 2023 et de 10 % en 2027. De l'avis de l'ensemble des parties prenantes, ces objectifs sont déjà très ambitieux. Il ne semble donc pas pertinent de les relever.

privilégier dans le développement de la consigne, et le décret fixant la trajectoire de mise sur le marché d'emballages réemployés en verre, prévu par l'article 12, n'interviendra qu'après cette évaluation.

perdre du temps et de l'énergie à réemployer ces bouteilles ? En réalité, de nombreuses études démontrent l'intérêt environnemental du réemploi. L'impact environnemental des dispositifs de réemploi dépend de plusieurs facteurs, les principaux étant le taux de réutilisation du contenant,

les impacts provenant très majoritairement de la production du verre. Ainsi, une bouteille en verre réemployée a un meilleur bilan environnemental qu'une bouteille en verre recyclée dès les premières réutilisations. Une étude de l'Ademe de 2018 a analysé dix dispositifs de réemploi du verre. Elle conclut que, sur tous les indicateurs et dispositifs étudiés, le système avec réemploi a une performance environnementale supérieure ou égale au système sans réutilisation.

j'invite mes collègues à voter l'amendement de Daniel Laurent, mais cela dans un esprit constructif,

Cet amendement vise à prendre en compte l'essor de la restauration à emporter ou livrée, essor qui a été accentué par la crise sanitaire. Il vise à préciser que les études de l'observatoire du réemploi et de la réutilisation, nécessaires à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique, devront également se pencher spécifiquement sur ce secteur qui a ses propres spécificités.

l'amendement n° 155. La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs, mais elle a besoin d'être soutenue. Allant dans le sens de la Convention citoyenne, nous proposons, comme nous l'avions fait lors de la discussion du projet de loi AGEC, la généralisation de la consigne du verre pour les cafés, hôtels et restaurants à l'horizon de 2023. Je vous rappelle que le Sénat avait à l'époque changé d'avis à la demande de la ministre : l'amendement avait d'abord été adopté, adopté, mais une seconde délibération l'avait rejeté ... Voilà une nouvelle chance de pouvoir avancer sur ce sujet ! La consignation en vue du réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels et restaurants. Les circuits logistiques de livraison, notamment pour

Cet amendement a pour objet de rendre à nouveau obligatoire l'usage d'emballages réemplissables consignés pour la bière, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels et restaurants. Les modalités d'application de cette obligation qui pourra être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, seront précisées par décret.

reviendrait plutôt à ces derniers d'organiser la consigne au service des cafés, hôtels et restaurants. Ensuite, une approche uniforme qui s'appliquerait à toutes les consommations dans ces lieux ne permettrait pas de tenir compte des particularités de chaque secteur.

pour les emballages du secteur des cafés, hôtels et restaurants et un financement spécifique par les éco-organismes de ces filières pour le développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages. C'est pourquoi je suis défavorable à ces amendements

n° 301 rectifié. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a introduit le dispositif de consigne, qui devait être généralisé sous réserve des résultats des bilans annuels, publiés par l'Ademe, évaluant ses impacts économiques et environnementaux. Ces bilans doivent permettre au Gouvernement de trancher sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de consigne obligatoire pour atteindre les objectifs de prévention et de gestion des déchets que la France s'est fixés. Cependant, ces bilans sont réalisés selon une approche nationale, et non territoriale, alors que la gestion des déchets relève par nature d'une gestion très locale et que l'impact environnemental de la consigne peut diverger selon les territoires. Par ailleurs, les résultats de ces études dépendent également de la typologie et du gisement des déchets concernés, tels que le verre ou le plastique. Le présent amendement a donc pour objet de territorialiser le dispositif de la consigne et de différencier sa mise en oeuvre en fonction des différents gisements de déchets.

Il nous semble particulièrement nécessaire d'appréhender correctement la performance de la gestion des déchets- cela devrait être une priorité. Un dispositif à même de prendre en compte de manière plus spécifique la situation locale permettrait de nous rapprocher de nos objectifs de recyclage des déchets, notamment des déchets plastiques. Bien évidemment, des moyens importants sont déjà mis en place aujourd'hui, mais nous estimons qu'un bilan seulement national ne permet pas de répondre au mieux aux besoins de nos territoires. De plus, dès 2023, le Gouvernement pourra définir des modalités de mise en oeuvre pour le recyclage et le réemploi des bouteilles plastiques.

Nous le savons tous ici, le service public de gestion des déchets est, par nature, local et répond à des demandes qui diffèrent selon les municipalités, les intercommunalités, les départements, voire les régions.

Comme toujours, agir efficacement et surtout intelligemment demande de se placer au plus près du terrain.

Le service public de gestion des déchets est, par nature, local ; il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisements. De la même manière, une généralisation de la consigne n'a aucun sens sur l'ensemble du territoire. Son déploiement doit être réalisé uniquement dans les zones qui n'atteignent pas les performances cibles. Le présent amendement vise à apporter cette dimension locale, qui est nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu pour laisser la place aux emballages plastiques, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, le réemploi des emballages entraîne un gain environnemental indiscutable, en évitant l'extraction de nouvelles ressources et en diminuant le nombre d'emballages à recycler, incinérer ou enfouir. Souhaitée par 88 % des Français selon une enquête de l'Ademe, la réintroduction du système de consigne pour réemploi sur les emballages en verre fut l'une des propositions des membres de la Convention citoyenne pour le climat. Adossée aux travaux de l'observatoire national du réemploi et de la réutilisation, cette généralisation de la consigne s'effectuera progressivement et en lien avec les différentes parties prenantes, pour être effective en 2025. Instaurer un cadre juridique opérationnel pour la reprise des emballages, comme tend à le faire cet amendement, permettra d'assurer le succès des systèmes de consigne à travers une incitation financière claire pour les consommateurs.

l'obligation de mettre en place une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu'ils soient lavables et réutilisables, pourra être généralisée, et cette généralisation n'entrera pas en vigueur avant le 1 janvier 2025. Fini donc le calendrier échelonné Certes, les travaux en commission ont permis de redonner de la couleur à cet article : l'amendement qu'elle a adopté a ainsi pour objet qu'une évaluation des dispositifs de consigne aux fins de réemploi pour les emballages en verre devra être menée avant le 1 janvier 2023 par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation. C'est le retour d'une échéance ... Cet amendement visait par ailleurs à compléter l'article L. 541-1 du code de l'environnement, afin que le décret définissant la proportion proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France détermine plus spécifiquement une trajectoire d'évolution, soit des obligations réelles. Le réemploi d'une bouteille en verre entraîne, nous le savons, 85 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à son équivalent à usage unique, 57 % par rapport à son équivalent en aluminium et 70 % au regard de son équivalent en plastique. Voilà autant d'arguments qui plaident en faveur de la généralisation de la consigne du verre à l'horizon de 2025, comme tend à le faire cet amendement. L'amendement

aurait pu être très touchant, mais ce sont les mêmes industriels qui, après avoir utilisé pendant des années un système de consigne parfaitement efficace, ont décidé de basculer vers des emballages jetables par seul souci de rentabilité. ont alors avancé une idée très simple : miser sur la responsabilité du consommateur pour cacher leur propre irresponsabilité. Néanmoins, nous savons aujourd'hui que la consigne pour réemploi doit être largement favorisée par rapport au recyclage d'emballages à usage unique. En outre, la consigne pour réemploi et réutilisation est une pratique à laquelle l'immense majorité des consommateurs est favorable : d'après une enquête de l'Ademe, 88 % d'entre eux trouveraient utile de disposer dans leurs magasins de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi et réutilisation.

L'article 12 propose une expérimentation- nous en avons parlé -et nous saluons les apports de la commission pour la densifier. Cependant, nous pensons qu'il est indispensable d'aller plus loin. Le présent amendement, qui a été travaillé avec de nombreuses ONG, notamment Zero Waste France, a donc pour objet de rétablir en France la pratique historique de la consigne pour les emballages en verre à partir de 2025. La date nous semble tout à fait raisonnable, et nous avons montré le chemin avec plusieurs amendements qui visaient notamment les centrales de lavage, la standardisation des contenants

Nadège Havet. L'option d'une transformation du Conseil national des déchets a été retenue ; l'objectif est de faire émerger une nouvelle instance de concertation dédiée à l'économie circulaire. Le décret est paru le 9 juin dernier le Conseil national de l'économie circulaire sera cette nouvelle enceinte destinée à traiter, outre les questions relatives aux déchets, déjà suivies par le Conseil national des déchets, les sujets de consommation et de production durables, notamment les sujets d'allongement de durée de vie des produits par le recours au réemploi, à la réutilisation et à la réparation, d'approvisionnement durable ou de lutte contre le gaspillage des produits. À présent, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie auront la possibilité de saisir pour avis cette instance consultative sur toutes les questions relatives à l'économie circulaire, de l'extraction des matières à la gestion des déchets, hormis les déchets radioactifs. Le Conseil pourra également s'autosaisir de toute question d'intérêt national concernant l'économie circulaire.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement repose sur une logique assez simple : il s'agit d'inciter aux bonnes pratiques environnementales et de décourager les mauvaises, ce qui est la logique même des filières de responsabilité élargie du producteur, Malheureusement, les industriels qui produisent des déchets qui ne sont pas valorisables et qui ne s'inscrivent pas dans une filière de responsabilité élargie du producteur ne paient aucune écocontribution et ne participent donc en rien à la gestion de ces déchets. Les entreprises les plus polluantes sont donc avantagées par rapport à celles qui sont soumises à une REP ; il s'agit d'une forme de prime au cancre. Sans aucune participation de ces entreprises polluantes à la gestion de leurs propres déchets, c'est aux collectivités de supporter entièrement le coût de cette gestion, et c'est également à elles qu'il revient de s'acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes que les collectivités doivent payer pour chaque tonne de déchets enfouis ou incinérés. Comment est-il possible, dans cette situation, de développer notre capacité de gestion des déchets, de réduire le volume de déchets stockés et d'éviter l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, augmentation qui se répercutera automatiquement sur le contribuable ? Par ailleurs, comme vous l'avez souligné, madame la ministre, il est important que les propositions de nos concitoyens viennent enrichir notre travail parlementaire, et cet amendement tend à s'inspirer de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d'emballage.

Cet amendement vise à s'attaquer à certains produits emblématiques, selon nous, de notre modèle de consommation de plastiques à usage unique. Il s'agit d'interdire la mise sur le marché de bouteilles d'eau en plastique de moins de 50 centilitres- en somme, nous interdisons les contenants plastiques de 20 ou 33 Il faut rappeler certains chiffres effrayants : quelque 25 millions de bouteilles en plastique sont consommées, puis jetées chaque jour en France, et moins de la moitié est ensuite recyclée. Ce type de petits contenants nous semble en totale contradiction avec les objectifs de l'économie circulaire et de la préservation de l'environnement. Nous avions proposé un amendement similaire il y a deux ans, lors de l'examen du projet de loi AGEC, et il nous avait été répondu qu'il fallait se donner le temps de la réflexion, notamment pour les industries qui sont affectées.

loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, dite loi AGEC, a élargi aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n'avaient plus l'usage aux organismes agissant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. Auparavant, cette possibilité n'était ouverte qu'à l'État et à ses établissements publics. Cette loi n'introduit aucune distinction entre les organismes à but commercial lucratif et ceux qui sont à but non lucratif, ce qui freine les activités commerciales des recycleries culturelles à but non lucratif et risque de conduire au gaspillage d'une partie des rebuts issus des établissements publics. cet amendement, nous proposons donc d'ouvrir les catégories de bénéficiaires aux professionnels de la recyclerie culturelle ayant les possibilités effectives de traiter l'intégralité des volumes de matériaux issus du secteur culturel public. Cette mesure permettrait de développer des emplois, de réduire sensiblement la quantité de déchets produits et de soutenir le secteur culturel, durement touché par la crise sanitaire. La parole est à Mme Martine

gratuitement les biens de scénographie dont ils n'avaient plus l'usage aux organismes agissant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. Précédemment, cette possibilité n'était ouverte qu'à l'État et à ses établissements publics. Néanmoins, alors que la loi exclut, à juste titre, les organismes à but commercial lucratif, elle n'introduit aucune distinction avec les organismes à but commercial non lucratif, qui utilisent les bénéfices de leur activité commerciale au service de l'intérêt général et non en vue de susciter un profit. Cette particularité freine les activités commerciales des recycleries culturelles à but non lucratif. Leur modèle économique repose pourtant sur l'investissement des bénéfices pour soutenir la culture dans sa transition vers l'économie circulaire et le réemploi. À titre d'exemple, pour la seule année 2020, La Réserve des arts a collecté 700 tonnes de rebuts, pour un taux de réemploi de 90 %, ce qui a permis de fournir des matériaux vendus à prix solidaire pour ses 8 000 adhérents. Restreindre l'accès du dispositif de cession aux organismes à but non commercial risque de conduire au gaspillage d'une partie des rebuts issus des établissements publics. Il est donc nécessaire d'ouvrir les catégories de bénéficiaires aux professionnels de la recyclerie culturelle ayant les possibilités effectives de traiter l'intégralité des volumes de matériaux issus du secteur culturel. Lever ce frein à la collecte de biens de scénographie est de nature à vivifier un secteur durement touché par la crise sanitaire, en prévision de la réouverture et de la reprise de la vie culturelle partout sur le territoire.

intervenant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable à recevoir des dons de biens de scénographie dont l'État et ses établissements publics, ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'ont plus l'usage. Il vise également à autoriser la cession de ces biens à titre onéreux pour permettre aux recycleries culturelles à but non lucratif de recevoir ces dons. Ces recycleries permettent de valoriser une part très importante des matériaux réemployables par les professionnels de la culture et de la création. À titre d'exemple, selon l'association La Réserve des arts, cette mesure permettra de développer 1 000 emplois sur la filière du réemploi des biens de scénographie dans les trois ans sur tous les territoires, de réduire d'environ 5 millions de tonnes par an la quantité de déchets produits en permettant aux recycleries culturelles de mettre en oeuvre des activités de réemploi et de réutilisation auprès des structures culturelles nationales, mais également de soutenir 271 000 professionnels du secteur culturel en leur donnant accès à des matériaux à tarif solidaire, les soutenant ainsi dans leurs productions.

Dans le cadre de la loi AGEC, les sénateurs de notre groupe ont fait adopter un amendement ayant pour objet la remise d'un rapport sur la question essentielle de l'obsolescence logicielle et sur la nécessité de réfléchir à des mesures visant à allonger la durée de vie des produits.

Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de recycleries, de ressourceries ou encore de points de collecte d'associations caritatives. Ces structures se développent et ont déjà un impact significatif sur notre gestion des déchets, avec plus de 200 000 tonnes de déchets réemployés ou recyclés, soit plus de 400 tonnes annuelles par structure, selon les chiffres de l'Ademe de 2017. Nous attendons leur mise à jour grâce au nouvel observatoire du réemploi. La pratique du réemploi, en plus d'être particulièrement vertueuse d'un point de vue écologique, est créatrice d'emplois et de lien social ; c'est un vecteur d'éducation populaire et de dynamisme local. Chaque élu ayant vu naître une ressourcerie sur son territoire peut mesurer l'ensemble des bénéfices qu'elle apporte aux communautés locales. Seulement, pour avoir un impact national, le réseau d'équipements de réemploi doit fortement se densifier. En cohérence avec la compétence déchets, nous proposons de mettre en place au moins un équipement par EPCI, et, pour faire face aux volumes, qui peuvent rapidement devenir considérables, au moins un par tranche de 22 000 habitants en zone urbaine. Ces 2 500 ou 3 000 nouveaux équipements permettraient d'employer des dizaines de milliers de personnes et de réutiliser ou valoriser des centaines de milliers de tonnes de déchets. Cela réduirait également la pression sur nos déchetteries, dont le maillage est d'une pour 14 000 habitants.

La fixation d'un objectif si précis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qui pose les grands principes et objectifs de la politique nationale de l'économie circulaire, ne me semble pas opportune. Je note toutefois que l'amendement est déjà satisfait par les amendements adoptés en commission à l'article 12 à renforcer le financement et la planification du déploiement des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment les laveuses et lieux de stockage des emballages consignés. L'avis de la commission est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

Pour commencer, nous proposons d'agir sur une pièce maîtresse des équipements électriques et électroniques, à savoir la batterie. Cet élément a une double caractéristique : il est à la fois une pièce indispensable et une pièce d'usure. Notons également que sa production requiert des techniques de production, ainsi que d'extraction de matériaux, qui sont très polluantes.

l'émergence, depuis plusieurs années, d'une pratique particulièrement détestable et anti-écologique : la soudure des batteries au châssis même des téléphones, qui interdit de fait tout remplacement de batterie par l'utilisateur et force donc ce dernier à remplacer son téléphone dès lors qu'elle est usée. Cette pratique, que l'on peut sans aucun sans aucun souci qualifier d'obsolescence programmée, doit être combattue par la loi. Voilà pourquoi nous proposons d'acter dans le code de la consommation ce principe de libre accès de l'utilisateur à la batterie, celle-ci devant être facilement détachable. Nous demandons également que la batterie, qui redevient ainsi une pièce remplaçable, soit mise à disposition en tant que pièce de rechange par le fabricant pendant une durée

est l'avis du Gouvernement ? Il s'agit d'amendements qui visent, d'un côté, à rendre les batteries de tout type d'appareil facilement accessibles afin d'être remplacées, et, de l'autre, à prévoir une durée de disponibilité des batteries de dix ans à compter de la fin de la commercialisation du produit. Sur le premier point, rendre obligatoire la possibilité d'accès aux batteries constitue une mesure relevant de l'écoconception des produits, qui est soumise à des règles harmonisées au niveau européen. Or un projet de règlement, en ce moment moment soumis à consultation par la Commission européenne, comporte une disposition en ce sens. Il fait l'objet de nombreuses négociations actuellement. Sur le second point, les batteries des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans, des moniteurs, des vélos à assistance électrique, des équipements de déplacement personnel motorisés constituent des pièces détachées de ces produits et sont donc déjà couvertes par une obligation de disponibilité d'une durée minimale de cinq ans après la fin de la commercialisation de ces produits, obligation qui est issue de la loi AGEC et du présent projet de loi. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur ces amendements, qui sont satisfaits.

à M. Guillaume Gontard. Lorsqu'un produit électroménager ou un produit électronique tombe en panne, l'absence de pièces détachées rend sa réparation difficile, voire impossible, si le fournisseur d'origine était le seul à posséder ces pièces détachées.

d'abord, nous souhaitons augmenter la durée de disponibilité des pièces détachées, que nous fixons ici à quinze ans pour l'électroménager et à dix ans pour l'électronique. Ensuite, nous voulons favoriser l'utilisation par les fabricants et les réparateurs agréés de pièces détachées issues de l'économie circulaire, et ce afin d'accroître la disponibilité des pièces. Enfin, lorsqu'une pièce détachée n'est plus mise à disposition par le fabricant, ce dernier devra rendre disponible le plan 3D de la pièce. D'autres fabricants, ou même certains particuliers en possession d'une imprimante 3D, par exemple, pourraient ainsi reproduire les pièces détachées qui ne sont plus fournies par le fournisseur d'origine. La loi prévoit une disposition analogue, mais les règles relatives à la propriété actuelle la rendent souvent difficilement applicable. Cet amendement, s'il était voté, compléterait opportunément ce que nous avons adopté dans la loi AGEC. est à M. André Guiol. Cet amendement tend à modifier l'article L. 111-4 du code de la consommation, dans la rédaction qui entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2022, afin de renforcer l'obligation des producteurs en matière de disponibilité des pièces détachées pour tout bien matériel fabriqué ou importé en France. de porter de cinq ans à dix ans la durée minimale de mise à disposition des pièces détachées des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, d'écrans et de moniteurs. Ensuite, il vise la possibilité de mettre à la disposition des vendeurs professionnels ou des réparateurs, qu'ils soient agréés ou non, des pièces détachées issues de l'économie circulaire pour certaines catégories définies par décret. L'amendement

L'obsolescence programmée et l'évolution technique des matériaux des cycles pèsent sur la durée de vie potentielle des vélos, alors que, selon l'Ademe, ces derniers ont un potentiel de réemployabilité très fort, à plus de 80 %. 80 %. Le présent amendement vise à lutter contre l'obsolescence programmée, qui met à mal l'un des piliers de la transition écologique, c'est-à-dire le principe des mobilités douces, en fixant la disponibilité minimale des pièces détachées et des outillages correspondants à quinze ans minimum. La disponibilité des pièces détachées sur la durée de vie d'un produit n'est utile, bien sûr, que si l'outillage nécessaire à leur installation est également disponible. Or les producteurs recourent de plus en plus à de l'outillage non universel. donc pour objet d'inscrire dans la loi une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et de l'outillage pour les cycles, se fondant sur leur durée de disponibilité moyenne actuelle. Cette durée est supérieure à la durée de vie moyenne des vélos, et le potentiel de réemployabilité technique des vélos est élevé- 80 %, selon l'étude de préfiguration de la filière REP-ASL, de 80 % -, et 30 % du parc des cycles sont inutilisés, ce qui augmente considérablement l'âge moyen des cycles traités par les opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Il est donc nécessaire d'assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d'allonger encore cette dernière. La longévité exceptionnelle de ces produits est remise en question par la forte évolution tactique du matériel observée ces dernières années. Ainsi, une disponibilité minimale fixée à quinze dans la loi permettrait aux cycles d'être réparables sur une durée conforme à l'existant, d'éviter le risque d'un effet d'aubaine pour les metteurs en marché et de lutter contre l'obsolescence marketing. L'amendement n° 1445, présenté

les dix ans. Nous proposons une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et des outillages spécifiques pour la réparation des vélos. Ce type de produit se caractérise par sa longévité exemplaire. Il arrive régulièrement que les ateliers de réparation redonnent vie à des vélos parfois très anciens. Or il se trouve que certaines pièces détachées sont indisponibles en raison d'une obsolescence technique. Le potentiel de réemployabilité des vélos est élevé- plus de 80 % -, et 30 % du parc des cycles sont inutilisés, ce qui augmente considérablement l'âge moyen des cycles traités par les opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Il est donc nécessaire d'assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d'allonger encore cette dernière. C'est pour cette raison que nous proposons une durée supplémentaire minimale de huit ans. est l'avis de la commission ? La durée de disponibilité peut déjà être augmentée au-delà des cinq ans par voie réglementaire, lorsque la durée de vie moyenne des produits le justifie. Il ne me semble donc pas opportun de fixer une durée législative de huit ans, dix ans ou quinze ans, qui pourrait poser un certain nombre de difficultés,

est à M. Hervé Gillé. Nous proposons de renforcer l'information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées avant l'achat d'un bien. Actuellement, cette information n'est rendue obligatoire que dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l'information aux distributeurs. La loi ne prévoit pas d'obligation d'information négative. Ainsi, un fabricant qui ne propose pas de pièces détachées n'a aucune obligation de le signaler, tandis qu'un fabricant qui fait l'effort d'afficher la disponibilité des pièces détachées pourra se voir sanctionné s'il ne parvient pas à les fournir. Notre proposition relève donc du bon sens. Le consommateur doit être informé lorsque les pièces détachées sont disponibles, mais également lorsqu'elles ne le sont pas. En renforçant l'information sur la réparabilité des produits, on oriente mieux le consommateur vers une consommation durable et responsable.

de limiter les renouvellements en terminaux neufs des utilisateurs, et, troisièmement, d'encourager la filière du réemploi et du reconditionné, source d'emplois peu délocalisables bénéficiant aux territoires. Pour ce faire, il convient d'inciter les utilisateurs à retourner leurs appareils en magasin lorsqu'ils ne les utilisent plus, au moyen d'un système de consigne versée lors de l'achat d'un appareil neuf et remboursée lors du retour dudit appareil en magasin. mesure incitera les utilisateurs à ne pas conserver d'appareils fonctionnels inusités. En outre, elle dynamisera les filières nationales de réemploi, en mettant des stocks dormants sur le marché et en faisant participer les professionnels de manière plus massive qu'actuellement. Ces derniers évolueront ainsi vers une prise en compte plus importante du réemploi et du reconditionné dans leur modèle économique.

de gaz à effet de serre. Il s'agit ici d'un domaine sur lequel nous pouvons et devons agir. Le Sénat l'a bien compris en votant plusieurs dispositions de la proposition de loi sur l'empreinte environnementale du numérique qui vont dans ce sens. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller encore plus loin.

ces appareils contiennent des ressources, des terres rares, qui pourraient être réutilisées. Nous vous proposons ainsi d'acter un principe simple : les vendeurs de téléphones doivent proposer aux consommateurs soit une consigne au montant proportionnel

Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire.

du fait du secret industriel, de la dilution des responsabilités et des moyens juridiques dont dispose le secteur privé. Dès lors, si la loi ne fonctionne pas, il faut changer la loi ! Nous proposons donc, en lien avec le combat que mènent actuellement nos collègues écologistes au Parlement européen, de remplacer le délit d'obsolescence programmée par un délit d'obsolescence prématurée. Nous vous proposons de définir celle-ci

amendement, nos collègues écologistes pointent une problématique réelle, celle de l'obsolescence non pas programmée, mais prématurée.

Deuxièmement, on est bien face à une malfaçon et à une entreprise récalcitrante : ce n'est qu'à la suite d'une action de groupe aux États-Unis, puis d'une action coordonnée par l'UFC-Que choisir et d'autres associations de consommateurs en Europe, afin d'alerter la Commission européenne, que Nintendo a commencé à admettre l'existence d'un problème. À l'heure actuelle, il n'est toujours pas question d'un remplacement gracieux des matériels défectueux une fois la garantie expirée, et cela malgré l'absence totale de lien entre l'utilisation des périphériques et leurs dysfonctionnements. Les données du problème sont finalement assez simples : on estime que, dans 60 % des cas, la défaillance des manettes Joy-Con a lieu quelques semaines

Pour autant, une disposition utile ne doit pas se transformer en casse-tête pour les entreprises : cela ne profiterait à personne. L'objet de cet amendement est donc tout simplement de mettre en oeuvre un délai raisonnable, pour que la filière puisse se mettre en ordre de marche.

améliorer la mise en oeuvre du dispositif, en permettant de déterminer par voie réglementaire, pour chaque catégorie d'équipement concernée, un délai d'application qui soit pertinent et réaliste. Cela nous aiderait beaucoup dans la mise en oeuvre de la loi AGEC. Je mets aux

Bigot. Cet amendement vise à inscrire, au sein de la liste des filières mentionnées comme étant prioritaires pour la création d'un fonds de réemploi, la filière à responsabilité élargie des producteurs, ou filière REP, dédiée aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

Il n'est pas envisageable aujourd'hui de mettre en place une filière REP dans le secteur de la construction du bâtiment sans considérer la place du réemploi dans cette même filière. La création d'un fonds de réemploi au sein de cette filière REP permettra de soutenir l'ensemble des projets qui existent ou émergent, ce qui contribuera au déploiement de cette filière innovante et pleine d'avenir, au plus près des besoins des territoires.

L'affichage obligatoire d'un indice de réparabilité permet d'informer les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des équipements électriques et électroniques. Cette information a pour objet principal d'orienter les consommateurs vers des comportements d'achat de produits plus facilement réparables. cet indice deviendra un indice de durabilité, notamment par l'ajout de nouveaux critères, comme la robustesse ou la fiabilité des produits. Pour donner plus d'efficacité au dispositif, cet indice serait également susceptible de servir de référentiel pour les producteurs, les importateurs et les distributeurs, qui pourraient ainsi anticiper une interdiction de mise sur le marché des produits dont l'indice de durabilité serait inférieur à un seuil fixé par décret. Il est proposé que cette interdiction entre en vigueur au 1 janvier 2025.

que pour la lutte contre le changement climatique. En effet, il est extrêmement dommageable pour la planète et pour le porte-monnaie de nos concitoyens que la défaillance d'une seule pièce impose le remplacement d'un appareil Selon l'Ademe, chaque Français jette tous les ans plus de 15 kilogrammes de matériel électrique et électronique, pour en racheter 23 kilogrammes, soit presque 90 millions d'appareils. Il y a donc une véritable inflation en la matière, alors même qu'une grande partie de ces appareils reste largement utilisable. Heureusement, Éco-systèmes parvient à recycler près des trois quarts de ces objets, mais c'est vite oublier que l'on estime qu'environ un tiers des appareils jetés échappe à cette initiative. L'indice de réparabilité est une option intéressante, dans la mesure où il permet aux futurs acheteurs de se projeter dans un usage long et de privilégier, à caractéristiques équivalentes, l'achat d'un appareil qu'ils pourront réparer. Néanmoins, ce n'est pas suffisant : quel intérêt a-t-on à se lancer dans une réparation si l'on doit faire importer les pièces ? Quel intérêt a-t-on à réparer son appareil si le prix d'une pièce neuve est presque le même que celui d'un nouvel appareil ? enfin, à prendre le risque d'aggraver la situation en endommageant une nouvelle pièce ? Il faut donc aujourd'hui aller plus loin et mettre en oeuvre une politique plus volontariste. Vous verrez que, si l'on interdit la mise sur le marché des produits dont l'indice de réparabilité est inférieur à 3 ou à 4, les fabricants parviendront très vite à proposer des appareils dont le seuil de réparabilité sera largement plus haut Restera problématique la situation des appareils qui font l'objet d'un monopole de fait, notamment en matière de périphériques, mais c'est bien ce genre d'actions qui permettra de renforcer la lutte contre le gaspillage.

l'amendement n° 7 rectifié . Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation doit comprendre un volet relatif à l'économie circulaire. La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d'activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l'attitude des consommateurs permettent de penser qu'une rupture vis-à-vis de notre modèle de production et de consommation